Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, dès le mois de juillet 2017, le Premier ministre était venu l'affirmer devant vous à l'occasion de sa déclaration de politique générale : la Nouvelle-Calédonie est une priorité pour le Gouvernement, et en particulier, bien sûr, pour le ministère des outre-mer.

Élaboré à l'issue du comité des signataires organisé au mois de novembre, soumis immédiatement à l'avis du Conseil d'État et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, avant son passage en conseil des ministres en décembre, il vous est présenté aujourd'hui.

qui vient solder une difficulté apparue il y a plusieurs années dans les discussions relatives aux listes électorales, l'ensemble des institutions de la République auront démontré leur pleine mobilisation pour contribuer, chacune dans ses compétences, à soutenir la Nouvelle-Calédonie, à lui permettre d'avancer. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, depuis trente ans, est celle d'un dépassement des antagonismes, des barrières culturelles et identitaires, pour ériger un modèle politique unique au monde. Ce modèle repose sur la conviction qu'il appartient à tous de contribuer au vivre ensemble et à la définition de ce que doit être le destin commun de celles et ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie. le plan politique, cela a conduit à élaborer un schéma institutionnel profondément original. Localement d'abord, avec une architecture en trois provinces, un congrès et un gouvernement. Surtout, dans l'esprit de l'accord de Nouméa, et afin de bâtir tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain, les membres de l'exécutif, élus à la proportionnelle, représentent toutes les tendances politiques. Majorité et opposition se côtoient au sein d'un collège dans lequel le consensus est au fondement de toutes les décisions. Le fait majoritaire, comme principe de décision collective, a donc subi des aménagements forts pour que la majorité tienne compte des intérêts des autres

La démocratie, c'est l'élection à la majorité. Mais la prise de décision majoritaire n'est pas le seul chemin que peut suivre la démocratie pour se déployer. Cette approche particulière de la prise de décision est à l'oeuvre avec le troisième partenaire des différents accords qu'est l'État. Lui aussi participe à la recherche permanente du compromis et du consensus. L'État est le garant des accords conclus. Il est le partenaire qui, avec ses moyens et son expertise, accompagne la réflexion collective, rappelle aussi les limites de ce que le droit permet. L'État est un acteur de la discussion : il l'anime, il propose des solutions, des idées, des compromis. C'est dans cet esprit que le Premier ministre a conduit les travaux du comité des signataires du mois de novembre dernier. Les échanges ont permis d'aboutir, vous le savez, à un compromis politique sur la question sensible de l'inscription d'office sur les listes électorales de personnes résidant en Nouvelle-Calédonie et répondant à différents critères leur permettant d'aspirer à participer au référendum. Le projet de loi organique qui vous est soumis transcrit cet accord politique fort. Il vise à garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin. Il a largement pris en compte les propositions émises par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, consulté à chaque étape sur l'ensemble des textes. Je tiens à le rappeler, car la confusion est parfois entretenue dans les esprits : le présent texte ne modifie pas le corps électoral,

les conditions pour participer au scrutin, avec comme finalité d'inscrire le maximum d'électeurs potentiels sur la liste électorale spéciale pour la consultation, la LESC. Environ 11 000 personnes, de statut civil coutumier ou de droit commun, sont potentiellement concernées par les nouvelles dispositions. Ce chiffre résulte de croisement de fichiers opéré

Pour inscrire ces personnes sur la liste électorale spéciale, une procédure d'inscription d'office sur la liste électorale générale était indispensable. L'avis du Conseil d'État, que le Gouvernement a consulté sur ce point, a permis de mettre en place une procédure adaptée. Outre les inscriptions d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale, le projet de loi organique ouvre la voie à la mise en place de bureaux de vote délocalisés, permettant aux électeurs des îles résidant à Nouméa de voter sur place. Cette disposition répond à une demande forte forte exprimée à plusieurs reprises par les élus de Nouvelle-Calédonie qui craignaient que des électeurs ne doivent renoncer à participer au scrutin, faute de place dans les avions ou de moyens de s'offrir un tel déplacement. En corollaire, parce que ce qui est privilégié est le vote personnel des électeurs, compte tenu de l'enjeu, un encadrement plus strict des procurations a été jugé pertinent par tous. Le dispositif de droit commun

Mais je reviens à mon propos sur les modalités particulières d'élaboration des décisions concernant la Nouvelle-Calédonie. Depuis trente ans, qu'observons-nous ? La procédure particulière d'élaboration de la décision publique à l'oeuvre en Nouvelle-Calédonie a fini par irriguer les institutions nationales. Depuis trente ans, le sujet est préservé des querelles politiciennes, des coups d'un jour, de tout ce qui pourrait en réalité déstabiliser le territoire. Il faut s'en féliciter. Chacun a pris la mesure de l'enjeu. Et chacun a pris conscience qu'il endosserait une responsabilité immense s'il ne s'inscrivait pas dans cette démarche engagée par d'illustres prédécesseurs. Cette démarche se veut respectueuse des opinions de chacun pour définir un chemin collectif qui réponde aux aspirations de tous. Pierre Frogier me pardonnera l'usage d'un concept qui lui est cher, mais j'ai envie de dire que les palabres océaniens et, avec eux, le respect, l'écoute, la prise en compte sincère de l'autre et de ses contraintes ont fini par faire école jusqu'à Paris. Au moins lorsqu'il s'agit de la Nouvelle-Calédonie ... À ce titre, je me félicite que le travail conduit par le Gouvernement sur ce projet de loi ait avancé sereinement, dans un échange constructif avec le Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat doivent en effet prendre toute leur part dans les réflexions en cours. C'est pourquoi il est important que vous ayez eu l'occasion, monsieur le rapporteur, de vous rendre en Nouvelle-Calédonie. La mission d'information de l'Assemblée nationale fera d'ailleurs de même la semaine prochaine. Je me félicite également des améliorations que vous avez introduites dans le projet de loi organique déposé par le Gouvernement. Indéniablement, à l'issue de son examen par la commission des lois, ce texte est mieux rédigé. Je pense en particulier à la réécriture d'une partie du premier article, qui y a gagné en clarté, à laquelle, je le sais, vous veillez. Je pense aussi à l'harmonisation des écritures entre les deux premiers articles.

contiendra des dispositions essentielles sur l'organisation de la campagne. Il fixera également les termes de la question posée. Le Gouvernement juge donc normal que le congrès, par dérogation aux principes habituels organisant les consultations, émette un avis. Le texte est mieux écrit, par conséquent moins susceptible d'être remis en cause. C'est essentiel. Le plus important, c'est que ce travail a été conduit dans le strict respect des équilibres fixés lors du comité des signataires. Les échanges informels entre nous ont également permis d'améliorer sensiblement la rédaction de l'amendement présenté par le Gouvernement concernant la répartition du temps de parole pour la campagne officielle, ainsi que les modalités d'intervention du CSA, Le sujet est important pour les partis politiques locaux. Je me permets de croire que les interrogations légitimes que vous avez soulevées ont été prises en considération et que des réponses auront pu y être apportées. Par ailleurs, le Gouvernement vous présentera un amendement visant à introduire le principe d'un remboursement plafonné des frais de campagne. C'est l'usage en matière de référendum. Un dispositif identique avait d'ailleurs été mis en place pour le référendum sur l'accord de Nouméa en 1998. C'est aussi un vecteur pour assurer une forme d'égalité entre les partis, qui ne disposent pas tous des mêmes moyens. Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de dire encore quelques mots sur la Nouvelle-Calédonie en guise de conclusion, au-delà du projet de loi dont nous allons entamer la discussion. ne résume pas, tant s'en faut, l'ensemble des actions conduites par le Gouvernement. La tâche importante que constitue la préparation de l'échéance référendaire suscite une mobilisation de l'ensemble des services de l'État. Ainsi, comme vous l'aviez souhaité, le ministère de la justice vient-il de désigner de désigner une dizaine de magistrats pour permettre aux commissions électorales de fonctionner. Nous travaillons également avec le ministère des affaires étrangères sur toutes les actions qui engagent les Nations unies.

anticipation de la mission d'observation sollicitée par les signataires pendant le scrutin. Surtout, la consultation n'est pas le seul horizon de notre action. L'État a réaffirmé son soutien à la Nouvelle-Calédonie dans le financement et la mise en oeuvre de politiques publiques essentielles. Une attention particulière a été portée aux crédits du budget opérationnel de programme, ou BOP 123, qui financent les contrats de développement et donc, concrètement, des investissements et des projets qui changent la vie quotidienne des Calédoniennes et des Calédoniens. Nous conduisons également, dans le cadre des assises des outre-mer, une réflexion collective, regroupant l'État, les institutions locales, les associations et tous les citoyens qui souhaitent y prendre part, sur la question spécifique de la jeunesse calédonienne.

et devraient -être le premier temps d'une mobilisation politique et sociétale en faveur de ceux qui sont la Nouvelle-Calédonie de demain et qui parfois, isolés, désocialisés, partent à la dérive. L'État a également souhaité que la Nouvelle-Calédonie, qui souffre de difficultés spécifiques pour ce qui concerne la sécurité, bénéficie d'un accompagnement dédié.

Le ministre de l'intérieur a confirmé, la semaine dernière, que Nouméa bénéficierait de l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien dans l'un de ses quartiers, avant- je le souhaite -un élargissement à l'ensemble de l'agglomération. À travers toutes ces actions s'exprime la conviction que le référendum est une étape dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais comme le Premier ministre l'avait dit au Sénat, en août dernier, la question qui sera posée ne porte pas sur le destin commun, qui doit continuer de se construire. La Nouvelle-Calédonie doit continuer d'avancer et de porter des projets et des ambitions. C'est pourquoi j'ai récemment rappelé la nécessité que, en parallèle de ces travaux préparatoires, se poursuive un dialogue politique, dont le Premier ministre a dessiné les contours lors de son déplacement à Nouméa. Il me semblait indispensable, avant de nous plonger dans la technicité de ce projet de loi organique, de le réaffirmer devant vous au nom du Gouvernement. La parole

de ce territoire, ne peut se faire sans être imprégné d'un sentiment de responsabilité.

prévu pour l'automne prochain est, sans aucun doute, une étape, mais il n'est pas la fin de l'histoire.

des coopérations qu'ils veulent développer. Il n'y a alors plus véritablement de destin commun, de même qu'il n'y en a plus avec un seul territoire français ayant choisi l'indépendance. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du scrutin de cette année de décider où ira la Nouvelle-Calédonie. Conscients de l'importance de cet enjeu, nous devons, au moment où il s'agit de déterminer la composition de la liste électorale permettant aux citoyens de Nouvelle-Calédonie de se prononcer sur l'avenir du territoire, être attentifs

C'était déjà l'enjeu de la loi organique de 2015, dont j'étais également le rapporteur et qui a permis l'inscription sur la liste électorale spéciale de nombreux Calédoniens, qui n'auraient pas forcément pris l'initiative de demander cette inscription. Nous avons inauguré cette politique d'inscription d'office il y a maintenant près de trois ans. Lors des entretiens de Matignon qui ont réuni, le 2 novembre dernier, tous les signataires ou leurs héritiers de l'accord de Nouméa de 1998, la décision a été prise d'aller plus loin dans le processus d'inscription d'office, afin de n'oublier personne. C'est l'objet du texte qui nous est présenté. Il prévoit tout d'abord, parce que c'est la condition pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale, que des inscriptions d'office pourront être faites sur la liste électorale générale pour tous les résidents de Nouvelle-Calédonie dont la résidence est ancienne d'au moins six mois. Cette première opération effectuée, le texte dont nous avons à discuter permet l'inscription d'office, sur la liste électorale spéciale, de Calédoniens dont le centre des intérêts matériels et moraux sera présumé du fait que, premièrement, ils seront natifs de Nouvelle-Calédonie et, deuxièmement, ils y auront résidé au moins trois ans.

Le texte y répond, autant qu'il peut le faire et sans aller au-delà de l'accord qui a été conclu entre les parties calédoniennes sous les auspices du Premier ministre le 2 novembre dernier il prévoit que la présomption de détention des intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'on y est né et y réside depuis au moins trois ans, est une présomption simple,

si elle n'est pas automatique, ne peut être refusée qu'en fonction des éléments fournis par l'État. Ces éléments proviennent d'un certain nombre de fichiers, le principal étant celui de l'organisme de sécurité sociale propre à la Nouvelle-Calédonie, lequel va pouvoir établir qu'une personne est résidente depuis au moins trois ans, tout simplement parce que des cotisations sociales auront été versées pendant cette période.

Je n'assurerais pas que toutes les parties calédoniennes font exactement la même interprétation de ce texte, mais je suis sûr qu'il correspond bien à leur volonté commune, avec sa force, mais aussi avec ses limites. Il me semble qu'il ne nous appartient pas de modifier l'équilibre de ce texte, car nous risquerions, si nous le faisions, de nous écarter de cet accord et de provoquer nous-mêmes

avec cette facilité offerte aux électeurs des îles, il est prévu de restreindre le recours aux procurations, dont on a observé

qui nous sépare du référendum d'autodétermination, dans des conditions qui évitent les tensions inutiles. Nous pouvons ainsi espérer que, quel qu'en soit le résultat, ce scrutin sera validé par toutes les forces calédoniennes. Encore faudra-t-il, au lendemain de cette consultation, savoir prendre les initiatives qui rassembleront les Calédoniens. Incontestablement, la République et son gouvernement auront un rôle majeur à jouer pour éclairer le chemin et permettre à tous les

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a trente ans, les accords de Matignon mettaient fin aux événements sanglants qui avaient endeuillé la Nouvelle-Calédonie de 1984 à 1988 et culminé lors du drame atroce d'Ouvéa. Trente ans ! C'est à la fois long et dérisoire à l'échelle de l'histoire de 165 ans entre l'État français et cet archipel. Le 24 septembre 1853, à Balade, la France de Napoléon III, qui cherchait alors une terre nouvelle, libre de toute occupation européenne, pour y fonder une colonie pénitentiaire, parvint à ses fins, en proclamant la Nouvelle-Calédonie colonie française. De la grande révolte des Kanaks de 1878 au massacre d'Ouvéa, comment effacer de notre mémoire le sang versé inutilement à des milliers de kilomètres de la France ? Comment, trente ans plus tard, oublier la grande leçon de fierté

Aujourd'hui, le groupe politique que je représente confirme toutes ses positions antérieures. Comme nous approuvions la loi organique de 1999, qui a traduit dans notre droit les dispositions de l'accord de Nouméa, nous approuverons aujourd'hui ce projet de loi organique, qui précise l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et qui marquerait- -la fin

nous veillerons à ce que toutes les parties soient respectées, en particulier les indépendantistes. La résistance de certains à l'idée même d'une indépendance et la menace d'une coupure totale en cas de victoire indépendantiste seraient contraires à la volonté de laisser aux Néo-Calédoniens le pouvoir de décider de leur avenir. En novembre dernier, lors d'une rencontre avec une délégation du parti anti-indépendantiste Le Rassemblement, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que, en cas d'indépendance, la Nouvelle-Calédonie serait pleinement responsable des compétences qui lui reviendraient. C'est une façon de fermer la porte à quelque solution d'indépendance-association que ce soit, ce qui nous satisfait », déclarait alors le leader de ce parti. comme l'affirme Sarah Mohamed-Gaillard, spécialiste de l'histoire de la France dans le Pacifique, si l'indépendance reste un objectif, le contexte de la décolonisation dans le monde a beaucoup évolué ; elle indique que « les indépendantistes veulent construire une indépendance pas seulement souveraine, mais viable, et s'en donner les moyens, notamment économiques. Certains d'entre eux sont moins fermés que dans les années 1970. » Aussi, la France n'a nul intérêt à se recroqueviller sur des solutions passéistes. Mes chers collègues, ne sous-estimons pas un ressentiment bien légitime des populations kanakes ! Ne sous-estimons pas non plus les inégalités prodigieuses entre une classe très dominante, qui a notamment bâti sa richesse sur l'or vert, et une classe de laissés-pour-compte dans l'extrême pauvreté ! Certes, la question identitaire est au coeur de ce projet, mais il paraît difficile de discuter de l'avenir du pays sans parler aux populations La Nouvelle-Calédonie est-elle prête pour être autonome sur le plan économique sans les aides de la métropole encore importantes aujourd'hui ? De son côté, la métropole aurait-elle encore quelques intérêts à garder un pied sur le territoire- nickel, paradis fiscal ... ? Ne va-t-on pas lâcher une dépendance politique pour une dépendance économique ? une dépendance économique ? Ces questions doivent être posées et des réponses adaptées apportées. N'oublions pas que, en cas de victoire du « non » cette année, l'accord de Nouméa prévoit l'organisation de deux autres scrutins similaires à deux ans d'intervalle. Potentiellement, les Néo-Calédoniens pourraient donc être amenés à se prononcer de nouveau en 2020 et 2022. D'ici là, il est du devoir et de la responsabilité de l'État français d'accompagner la Nouvelle-Calédonie et de créer les conditions d'un développement pérenne, notamment en prenant en compte les atouts de l'archipel pour faire face au défi de la dépendance, que ce soit grâce à la ressource du nickel ou aux économies verte et bleue qu'il est possible d'exploiter pour valoriser le patrimoine intrinsèque dans le cadre de partenariats et d'accords avec les territoires du bassin de l'océan Pacifique. Dans la limite de son nouveau rôle à l'issue du scrutin, l'État français devra continuer à contribuer à la lutte contre les inégalités, à aider les provinces les plus fragiles à gagner la bataille du développement et, à terme, à faire en sorte que les différentes communautés ne réfléchissent plus par rapport à la France. Aujourd'hui, au-delà du référendum qui se prépare- nous serons très attentifs au bon déroulement de la campagne qui le précédera -, il s'agit d'anticiper l'issue du scrutin pour que les tensions endormies ou apaisées sur l'archipel ne se réveillent pas, si le respect des communautés composant le territoire venait à faiblir. Finalement,

monsieur le président de la commission, mes chers collègues, en juillet 2013, j'étais intervenu dans le débat sur l'actualisation de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et je reconnaissais bien volontiers mon ignorance des réalités sociologiques, historiques et politiques de ce territoire. Depuis, je pense m'être un peu rattrapé, notamment en me rendant sur place dans le cadre d'une étude triennale sur le foncier menée par la délégation sénatoriale Je suis toujours convaincu que la spécificité du modèle calédonien depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 est sans équivalent. est, néanmoins, l'héritage d'une histoire complexe, marquée par de violents affrontements entre communautés autour de la question de l'accession à l'indépendance. La signature des accords de Matignon avait mis un terme à plusieurs années de tensions ayant atteint leur paroxysme lors de la tragédie de la grotte Ces accords ont été suivis par celui de Nouméa et par sa traduction juridique, la loi organique du 19 mars 1999, qui prévoyait des transferts progressifs de compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie et la tenue d'une consultation de de la population entre 2014 et 2018 pour décider de l'avenir institutionnel de cette collectivité. Ce moment est aujourd'hui arrivé, mais l'une des questions essentielles de l'organisation de la consultation, qui devrait avoir lieu en novembre prochain, repose sur la composition du corps électoral qui y participera. Il existe en Nouvelle-Calédonie trois listes électorales distinctes, selon les règles fixées par la loi organique précitée de 1999. La première, dite liste électorale générale, regroupe les électeurs participant aux élections nationales françaises. La deuxième, dite liste électorale spéciale, permet aux électeurs inscrits de participer à l'élection des assemblées délibérantes spécifiques de la Nouvelle-Calédonie.

doivent se trouver dans l'un des huit cas prévus à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999. C'est l'inscription sur cette troisième liste qui fait l'objet de difficultés. Aujourd'hui, environ 160 000 électeurs y sont inscrits, tandis qu'entre 10 000 et 22 000 personnes pourraient demander à y figurer, si elles étaient inscrites sur la liste électorale générale. Le 2 novembre dernier, sous l'égide du Premier ministre, le XVI comité des signataires de l'accord de Nouméa a trouvé un consensus sur les modalités d'organisation du référendum d'autodétermination. Le présent projet de loi organique est la traduction de cet accord politique. Il permettra d'inscrire d'office sur la liste électorale générale les électeurs qui n'y figurent pas et qui ont leur domicile réel dans une commune située en Nouvelle-Calédonie ou y habitent depuis six mois au moins, conformément au droit commun. au droit commun. Il permettra également de procéder à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et domiciliés de manière continue pendant trois ans, lesquels seront réputés y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, il prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes éloignées de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa, mais résidant sur la Grande-Terre, pourront voter à Nouméa dans des bureaux de vote communaux délocalisés. Enfin, il rendra possible l'ouverture d'une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, la présence sur cette liste étant également l'un des critères au titre duquel il est possible d'être inscrit sur la liste électorale spéciale. Ce texte, qui est d'une importance capitale pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, marque l'engagement pris par ce gouvernement d'honorer sa parole et de permettre la plus large représentation à cette consultation, afin qu'elle se déroule dans des conditions sereines et transparentes et que le résultat qui en découle se révèle par conséquent incontestable. Ce résultat, quel qu'il soit, ne devra pas opposer deux camps : celui du « oui » et celui du « non Il devra permettre de continuer la construction de cette communauté de destin des Calédoniens, chère aux élus de ce territoire, notamment mes collègues et amis, Pierre Frogier et Gérard Poadja. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera en faveur de ce projet de loi organique.

je suis très ému de m'adresser à vous aujourd'hui, parce que le projet de loi organique que nous examinons me donne l'occasion de vous parler de mon histoire et, au travers d'elle, de l'histoire du pays. Vous me connaissez sous le nom de Gérard Poadja.

Tous deux ont été engagés volontaires au sein du Bataillon du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle pas moins de 2 000 Calédoniens, dont un millier de Kanaks, ont participé à la défense du monde libre. Mon père était, ces cow-boys calédoniens qui, à l'époque, dans les années 1930 à 1950, conduisaient sur plusieurs centaines de kilomètres les troupeaux de bovins de la province Nord jusqu'à Nouméa, afin d'alimenter la capitale en viande. Il a ensuite été éleveur sur sa propriété. C'était la concrétisation d'un rêve, mais ce rêve s'est fracassé à partir de 1983-1984 sur ce que l'on appelle pudiquement chez nous « les événements notre cheptel a été abattu à coup de sabre et de tamioc ; nos champs ont été saccagés, nos barrières coupées, notre famille menacée. Nous avons dû abandonner notre propriété, comme beaucoup d'autres Calédoniens de toutes origines de la Grande-Terre et des îles. Nous avons dû le faire, parce que, à ce moment-là de l'histoire, nous n'étions pas, politiquement, du bon côté ; nous étions du côté de la France, de la République.

qui n'a pas souvent sa place dans les palais de la République, c'est parce que mon engagement pour que la Nouvelle-Calédonie demeure au sein de la République française est un engagement de longue date, dont ma famille a payé le prix dans sa chair et dans son sang. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant mon attachement viscéral à la paix ! Celle qui a été tissée depuis que deux hommes d'exception, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont su se serrer la main au lendemain du terrible drame d'Ouvéa. Cette paix qui, trente années durant, au travers des accords de Matignon et de Nouméa, nous a permis de bâtir un vivre ensemble calédonien, dans lequel chacun, quelle que soit son origine ethnique, a appris, au fil du temps, à comprendre l'autre Nous arrivons aujourd'hui au terme de cet accord. Une consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté doit être organisée au plus tard en novembre 2018. Cette consultation majeure pour l'avenir de notre pays aboutira à un résultat, dont ni la légitimité ni la sincérité ne doivent pouvoir être remises en cause. C'est pourquoi, lors du XVI comité des signataires de l'accord de Nouméa, les partenaires politiques se sont unanimement mis d'accord sur trois points majeurs sur les listes électorales générale et référendaire tous les natifs du pays, qu'ils soient kanaks ou non kanaks ; favoriser le vote personnel des électeurs, en créant des bureaux de vote décentralisés pour les inscrits des îles qui résident sur la Grande-Terre encadrer de manière plus rigoureuse le recours au vote par procuration. Chacun de ces engagements a été respecté et, autant que nécessaire, repris dans les amendements que j'ai moi-même présentés lors de la Pour autant, cette consultation sur l'accession du pays à la pleine souveraineté porte en elle un vice originel : elle réduit de manière frontale les Calédoniens à ce qui les oppose, avec les risques de tensions ethniques, politiques et sociales qui en découlent. Comment, dès lors, poursuivre l'oeuvre de réconciliation et de paix de ceux qui nous ont précédés, tout en respectant cette échéance prévue par l'accord de Nouméa ?

Une déclaration qui nous permettrait de sceller nos convergences sur le destin commun, afin d'assumer plus sereinement nos divergences sur l'avenir du pays lors de Une déclaration sur ce qui fait notre ciment, nos acquis de ces trente dernières années, parmi lesquels le processus de décolonisation et d'émancipation, les valeurs calédoniennes qui nous lient, des institutions singulières à l'échelle de la République, des mémoires heurtées devenues au fil du temps une mémoire commune, et tout ce qui fait que l'on se sent calédonien. Cette déclaration permettra ainsi d'affirmer ce qui nous rassemble avant de nous prononcer sur ce qui nous divise. C'est ainsi que nous pourrons maintenir ce que nous avons de plus cher dans notre pays : la paix Chers amis, chers collègues, celui qui s'exprime à la tribune est un Kanak, qui appartient à une civilisation millénaire. Il est calédonien, aussi, parce qu'il a décidé de partager son pays avec celles et ceux qui, depuis 165 ans, ont contribué à sa mise en valeur. Il est français, enfin, parce que la grande histoire du monde a voulu que ce soit la France qui, en 1853, prenne possession de cette petite île du Pacifique. ce Calédonien, ce Français aujourd'hui devant vous revendique toutes ces appartenances qu'une grande partie des Calédoniens a appris à conjuguer. Je souhaite plus que jamais que, au lendemain du référendum, nous soyons capables de continuer à les conjuguer, ensemble, dans la France et dans la paix. Comme l'a dit mon grand frère coutumier Élie Poigoune, leader indépendantiste historique, « la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un grand frère, et ce grand frère, c'est la France ». Vive la Nouvelle-Calédonie ! Vive la République ! Vive la France

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, rapporteur de ce projet de loi organique, mes chers collègues, il est difficile de prendre la parole après Gérard Poadja, qui a parlé avec son coeur de son histoire, de ce qu'il vit en Nouvelle-Calédonie. En ce qui me concerne, je dois au hasard de la décision du président de la commission des lois de se rendre en Nouvelle-Calédonie pour procéder à des auditions afin de s'assurer que le texte qui nous est proposé est bien conforme à ce que souhaite le peuple de Nouvelle-Calédonie

il appartient au Gouvernement de prendre la décision. Fort heureusement, vous avez accepté l'idée de la consultation préalable du congrès, ce qui est de bonne démocratie. L'organisation de ce référendum doit être totalement incontestable. Il est fondamental que nul ne puisse, au lendemain du scrutin, dire que les dés étaient pipés, que le scrutin n'a pas été bien organisé. le sens de la présence très forte de l'ONU ; c'est le sens également de la présence de magistrats, qui vont être chargés de contrôler les opérations ; c'est le sens aussi de la demande

qui n'est pas irréfragable, comme l'a rappelé le président Bas, que leur centre d'intérêts matériels et moraux se trouve bien en Nouvelle-Calédonie. Tout cela, comme il nous l'a été rappelé, doit être tout à fait conforme à l'accord de Nouméa, lequel stipulait que le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie serait restreint aux personnes établies depuis une certaine durée, c'est-à-dire à celles qui, effectivement,

Enfin, et c'est le sens de votre dernier amendement, il faut que la campagne électorale puisse s'organiser du mieux possible, ces débats, qui ont lieu depuis des années, devant pouvoir continuer sereinement. Après, que se passera-t-il ? aboutit à l'autodétermination, la France devra sans doute accompagner l'assemblée constituante, permettre de constituer cet État de Nouvelle-Calédonie, et voir quels sont les partenariats que nous pourrons nouer avec ce territoire. et nul ne peut aujourd'hui anticiper sur un tel scrutin, car cela serait la pire des choses, surtout dans cet hémicycle, si la Nouvelle-Calédonie choisit de rester dans la République,

mais, dans l'intervalle, si le référendum n'aboutit pas à l'autodétermination, il nous faudra bien travailler, sans doute aussi dans cet hémicycle et dans nos commissions, sur la pérennisation du statut particulier pour réussir cette phase.

à la manière, en quelque sorte, de vider le Parlement de sa substance, alors que l'on voit bien que, en démocratie, les élus ont un rôle fondamental. Sans les élus qui se rencontrent au congrès, sans les élus qui oeuvrent au consensus, sans cette capacité de travailler ensemble, malgré des désaccords, on ne réussira pas.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voilà près de trente ans maintenant, les accords Matignon-Oudinot mettaient fin à une période de tensions sévères entre la communauté kanake et la communauté européenne sur le territoire calédonien ans, et derrière nous déjà, une longue série de négociations vers l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ces accords Matignon-Oudinot avaient prévu un temps de réflexion de dix ans, période de développement supposée instaurer des garanties institutionnelles et économiques pour le peuple kanak, dans l'attente de sa prochaine indépendance. À l'issue de ces dix années, le 5 mai 1998, le Gouvernement a signé l'accord de Nouméa

exception de domaines clés comme la défense, la sécurité, la justice, ou encore la diplomatie, ce transfert de compétences a marqué la première étape d'une reconnaissance de l'autonomie du territoire calédonien. À Nouméa encore, gouvernement français et représentants kanaks s'étaient entendus sur l'échéance de 2018 pour l'organisation d'un référendum sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. projet de loi organique a pour objet d'apporter les modifications législatives nécessaires pour faciliter les opérations de vote lors de cette consultation favoriser l'inscription sur les listes électorales. Il vise notamment à mettre en place une procédure exceptionnelle d'inscription d'office sur les listes électorales générales des communes de la Nouvelle-Calédonie pour tous les électeurs, qui, n'étant pas déjà inscrits sur une liste électorale, ont leur domicile réel dans une commune de la Nouvelle-Calédonie ou y habitent depuis six mois au moins. Il prévoit d'inscrire d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale. Ce texte permettra également, s'il est adopté, aux électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa de voter à Nouméa pour ce scrutin. Enfin, il élargit la possibilité d'ouvrir une période complémentaire de révision des listes électorales l'année du scrutin et garantit la sécurité juridique de l'organisation de la consultation. des lois a enrichi ce projet de loi organique sans en modifier l'équilibre. En effet, deux nouvelles dispositions ont été insérées : l'une encadrant plus strictement le droit de vote par procuration ; l'autre précisant que le décret de convocation des électeurs est pris après consultation à la fois du congrès et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pour conclure, je dirai qu'il est primordial que ce processus de consultation référendaire se déroule le mieux possible. Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera en faveur de ce projet de loi organique, dont les dispositions ont été adoptées, il faut le souligner, à l'unanimité par la commission des lois du Sénat.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, président de la commission des lois, mes chers collègues, prévue par l'accord de Nouméa de 1998, la mise en oeuvre de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie nécessite de transcrire dans la loi organique du 19 mars 1999 le résultat de l'accord politique obtenu au sein du comité des signataires de l'accord de Nouméa, tenu le 2 novembre 2017. Le dépôt tardif du texte sur le bureau du Sénat introduit une importante contrainte temporelle avec laquelle nous devons composer, compte tenu du nombre important de mesures réglementaires à publier et des délais de recours à respecter avant l'expiration du délai prévu par l'accord, en novembre 2018. Le Conseil d'État n'a pas manqué de souligner, dans son avis du 30 novembre 2017, un calendrier particulièrement serré. Depuis 1998, les tensions se cristallisent essentiellement autour de la composition de la liste électorale spéciale rassemblant les électeurs habilités à prendre part à la consultation sur la pleine souveraineté, ses partisans dénonçant l'exclusion de près de 23 000 Kanaks sur 90 000 en âge de voter, soit une part non négligeable du corps électoral total de près de 160 000 personnes. C'est pourquoi nos collègues Gérard Poadja, Pierre Frogier, ainsi que les députés Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, plaident auprès des partenaires politiques locaux et de l'État la nécessité de procéder à l'inscription d'office de ces quelque 11 000 natifs du pays sur les listes électorales. La conciliation entre cette préoccupation et la nécessité de permettre aux nouveaux résidents français de prendre part à la vie démocratique explique la coexistence de trois listes électorales distinctes en Nouvelle-Calédonie. Conformément à la volonté exprimée lors du XVI comité des signataires de l'accord de Nouméa, le projet de loi organique soumis à notre examen comprend diverses mesures pour garantir la légitimité du scrutin et favoriser la plus large participation des « populations intéressées » à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, garantissant ainsi la sincérité de la consultation à venir. venir. Ce texte traduit par conséquent fidèlement la volonté commune des signataires de l'accord de Nouméa, des représentants des institutions calédoniennes et des formations politiques locales.

émanant du président de mon groupe, Jean-Claude Requier, concernant, d'une part, l'information des électeurs, que nous considérons nécessaire, sur les modalités d'exercice du droit d'option, afin de garantir la sincérité du scrutin, et, d'autre part, les meilleures conditions d'information des électeurs quant aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration. Sur ce point, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a émis le souhait, dans son avis du 23 novembre 2017, de voir préciser le vote par procuration. Je rappellerai, pour clore ce débat, que l'avis du Conseil d'État souligne une fois encore les lacunes de l'étude d'impact fournie par le Gouvernement concernant les mesures relatives au régime des procurations. Madame la ministre, sur le plan strictement législatif, votre projet de loi organique entre dans le cadre légal en vigueur. Pourtant, mon groupe attire l'attention du Gouvernement sur l'exercice même qui va se traduire concrètement par l'organisation de la consultation. Le président de la commission des lois, dont je salue l'engagement sur ce dossier,

Monsieur le président, vous avez souligné en commission des lois, le 7 février, que cette consultation comportait des risques pour la concorde civile en Nouvelle-Calédonie. Notre collègue Gérard Poadja, auditionné par cette même commission, indiquait également qu'une consultation mal préparée pourrait provoquer des tensions ethniques et politiques. Ainsi, en contribuant à rendre le résultat incontestable, les dispositions de ce projet de loi organique sont de nature à favoriser une consultation référendaire apaisée, ... Exactement ! ... certes, mais j'aimerais ajouter une autre préconisation, qui concerne le texte même de la question posée. Je me suis personnellement confronté pendant deux ans à certains élus de mon territoire, ... Lesquels ? ... dont la volonté, relayée par le Gouvernement, était de vouloir introduire par voie référendaire une modification du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Gouvernement a finalement fait le choix de reculer, mais la question posée était, de mon point de vue, extrêmement ambiguë. Loin de vouloir ouvrir une polémique avec le Gouvernement, j'insiste néanmoins sur l'impérieuse nécessité de faire en sorte que la question posée pour la Nouvelle-Calédonie soit claire et sans aucune ambiguïté. La réponse doit être oui ou non. La formulation de la question ne doit pas être l'occasion d'ouvrir un nouveau débat sur l'avenir institutionnel, sinon les efforts déployés pour rendre incontestable cette consultation voleraient en éclats, et nous risquerions d'ouvrir une crise politique majeure que ce territoire n'a pas le luxe de s'offrir aujourd'hui. Je sais combien le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des forces politiques seront vigilants sur ce point. Mais, ne nous y trompons pas, cette consultation ne réglera pas le sujet de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

En fait, ce qui se joue depuis quelques décennies en Nouvelle-Calédonie, c'est le vivre ensemble, que j'associe au troisième pilier de notre devise républicaine : la fraternité. Dans un contexte que nos collègues calédoniens pourraient mieux décrire que moi,

Nous ne prétendons pas avoir la solution, et je crois que, sur ce sujet, il appartient aux Calédoniens eux-mêmes de construire cette troisième voie du vivre ensemble. Or celle-ci ne passe pas seulement par la loi ; elle passe par l'intelligence collective, qui irrigue la Nouvelle-Calédonie, et qui s'est traduite voilà quelques minutes dans les propos de notre collègue Gérard Poadja, Kanak, Calédonien et Français.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, la France ou l'indépendance ? L'indépendance ou la France ? Tel est le choix que les Calédoniens auront à faire avant la fin de cette année. C'est dans ce contexte que nous sommes appelés aujourd'hui,

On ne peut que se réjouir, bien sûr, qu'un accord ait été trouvé sur la question délicate de la composition de la liste référendaire. Cela devrait contribuer à rendre ce scrutin incontestable.

car le caractère de cette consultation exige que chacune et chacun d'entre nous s'expriment personnellement. Le vote par procuration doit rester l'exception. Il y va de la sincérité de ce scrutin d'autodétermination. donc en faveur de ce texte. Voilà pour ce qui est de la préparation technique de cette consultation, mais l'essentiel n'est pas là.

car les mots ont un sens -, lors de la consultation d'autodétermination. Que le Premier ministre de la France fasse référence dans son discours à un peuple distinct du peuple français qui, de surcroît, serait souverain, et ce à quelques mois du scrutin d'autodétermination, ne peut pas être une maladresse. Une telle expression marque une orientation : inscrire d'ores et déjà la Nouvelle-Calédonie en marge de l'ensemble français donner des gages aux indépendantistes, que l'on sait pourtant minoritaires parmi les citoyens calédoniens. C'est la poursuite de l'ambiguïté à laquelle nous ont déjà habitués les gouvernements de François Hollande pendant cinq ans. Signe des temps, d'ailleurs, comme sous la majorité précédente, c'est toujours l'ancien directeur de cabinet de François Hollande, haut fonctionnaire d'une grande respectabilité par ailleurs, qui représente l'État en Nouvelle-Calédonie et qui préside à nos échanges, dans une continuité tranquille, par-delà les alternances. Cette ambiguïté, elle est partout dans la manière dont l'État aborde cette consultation. Ne nous y trompons pas,

acteur dont l'avis n'est pas connu, le seul qui refuse de s'engager dans ce débat, le seul qui ne veut pas dire ce qu'il veut, c'est l'État Comme s'il avait peur de dire que le fait que des centaines de milliers de Français pourraient quitter l'ensemble national ne lui est pas indifférent. Est-ce si difficile pour l'État de dire son attachement à une Nouvelle-Calédonie dans la France ? Au lieu de prononcer ces mots simples, madame la ministre, vous nous demandez de nous réunir à Nouméa- j'ai bien entendu vos propos lors des voeux que vous avez prononcés en votre ministère -pour poursuivre le dialogue politique. Qu'est-ce que cela veut dire ?

l'hypothèse d'une Nouvelle-Calédonie dans la France, mais aussi celle d'une Nouvelle-Calédonie indépendante. Mais je ne tomberai pas dans ce piège Je n'ai certainement pas reçu mandat de préparer, même sous forme d'hypothèse de travail, le scénario d'une Nouvelle-Calédonie indépendante ou associée à la France. Toute l'histoire du parti politique que je préside, toute mon histoire personnelle tendent à permettre à la Nouvelle-Calédonie de rester française. Et l'État, à quelques mois d'un référendum politiquement mal préparé -je le dis et le répète depuis tant d'années -, voudrait que je donne ma caution à cette démarche ... Mes chers collègues, je vous le dis très clairement : l'État n'a, par définition, aucune légitimité pour préparer l'indépendance, tout simplement parce que l'indépendance serait la fin du lien politique et juridique avec la France. Dans ces conditions, madame la ministre, je vous demande solennellement, devant la représentation nationale, de préciser le cadre politique des groupes de travail animés par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie. Préparons-nous aussi l'indépendance, ou une solution qui s'y apparenterait ? J'attends de votre part une réponse claire, pour permettre à chacun de se positionner en conscience : oui, l'État vous demande d'évoquer aussi l'hypothèse de l'indépendance ; ou non, l'État prépare la seule situation qui relève de sa compétence, le compétence, le maintien dans la France. Il ne devrait pas être difficile pour un responsable national de répondre à cette question aussi clairement que je la formule. S'il s'agit de préparer notre avenir dans la France, comme c'est la responsabilité première de l'État, dites-le, et je m'y engagerai de toutes mes forces. Mais s'il s'agit aussi de préparer l'hypothèse d'une indépendance, ou d'une indépendance-association, je vous combattrai résolument. Madame la ministre, la première qualité d'un responsable politique est la lucidité. Or la lucidité, c'est de constater, comme je l'ai fait, que le temps de la recherche d'un nouvel accord politique est derrière nous. Signataire des accords de Matignon, signataire de l'accord de Nouméa, j'ai tenté pendant près de dix ans- oui, dix ans -d'emprunter tous les chemins possibles, sans exception, pour empêcher qu'un référendum brutal et mal préparé ne vienne anéantir tout ce que nous avions patiemment construit. Depuis six ans,

parfois même de me combattre. C'est sa responsabilité, mais qu'il assume désormais ses ambiguïtés successives. Ce que je demande à l'État, tout simplement, car il le doit à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, c'est de la clarté à la veille de ce référendum. Cela m'amène à ma seconde question.

: celle que l'État ne propose aux suffrages des Calédoniens une question alambiquée, une question ambiguë. pouvez-vous me confirmer que votre intention est bien de demander aux Calédoniens s'ils souhaitent, ou non, le maintien dans la France, sans aller à la recherche de formulations susceptibles de biaiser l'expression de leur volonté ? si le temps de la recherche d'un nouvel accord est passé, la période qui nous sépare de la consultation ne peut pas être celle de l'ambiguïté

et Territoires. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Jean-Louis Lagourgue l'a rappelé avec des mots pleins de sens : la Nouvelle-Calédonie s'apprête à tourner une page décisive de son histoire. novembre prochain, trente ans après les accords de Matignon, vingt ans après celui de Nouméa, le référendum devra bien ouvrir une nouvelle étape pour construire l'avenir de ce territoire. La page, aujourd'hui encore blanche, devra alors s'écrire avec l'aide et la participation de tous. Quelle sera-t-elle ? Nul à cet instant ne le sait, mais, en raison des accords intervenus, le référendum est inéluctable. On peut comprendre- je l'avais écrit avant de l'entendre -que Pierre Frogier et d'autres auraient préféré l'éviter, en raison de son caractère binaire.

L'esprit qui avait inspiré Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou n'était pas au rendez-vous. On peut le regretter, mais il faut le constater. Dès lors, il fallait commencer par réussir cette consultation pour passer à l'étape suivante.

nous avons besoin d'eux pour avancer dans la direction dans laquelle nous voulons tous aller ensemble. Pour coconstruire et préserver l'équilibre fragile de ce référendum, un comité dit des signataires de l'accord de Nouméa s'est réuni régulièrement pendant deux décennies. Il a assuré, parfois difficilement, un dialogue continu entre l'ensemble des parties prenantes. Il faudra, demain, avoir soin de consolider, sous une forme ou sous une autre, cette instance de dialogue,

Des thématiques essentielles y sont abordées, comme l'économie liée au nickel ou la jeunesse calédonienne et les enjeux qu'elle représente. Le Sénat est très sensible à cette approche. Le président Larcher avait mis en place, dès novembre 2015, un groupe de contact, qui existe toujours, chargé de réfléchir de façon large à l'avenir

La parole est à M. Robert Laufoaulu, pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis pour discuter d'un projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie. C'est dire la place spéciale, unique et primordiale qu'occupe ce territoire. Nous tous, responsables politiques, sommes tendus vers l'objectif fixé : organiser dans l'harmonie et la concorde le référendum inscrit dans la loi organique de 1999. Les dirigeants calédoniens ont assumé avec conscience leur devoir, et la consultation se fera dans la transparence et la confiance. Je veux m'associer aux salutations adressées à cette haute conscience des responsabilités dont font preuve les Calédoniens aux moments cruciaux de leur histoire le pari de l'intelligence, avec leur grande capacité à se rassembler lorsque les circonstances l'exigent et à se projeter ensemble dans l'avenir. Je tiens à saluer aussi l'engagement de l'État, qui s'est mobilisé pour dégager, conjointement avec les responsables calédoniens, la route quelque peu chaotique du référendum. Le Premier ministre, en présidant le dernier comité des signataires et lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie l'an passé, s'est inscrit dans la lignée politique des visionnaires éclairés et vigilants du dossier calédonien. Notre rôle, en tant que parlementaires, est d'accompagner la volonté des Calédoniens de tenir le référendum dans les termes du consensus qu'ils ont encadré. Avec le souci d'améliorer, peut-être, mais toujours, en tout cas, dans le respect fidèle de leurs décisions. Les résultats de la consultation sont, de l'avis d'un grand nombre d'observateurs, connus d'avance et très certainement en défaveur de l'indépendance. était-il nécessaire d'en passer par cette étape, qui risque de raviver de mauvais souvenirs, de créer un sentiment d'humiliation chez certains, d'en tenter d'autres de retourner à la violence ? Le questionnement sur un autre accord ou sur la déclaration commune pour le patrimoine commun était tout à fait légitime. Ce sont des questions qui me viennent à l'esprit, à moi qui ai connu, vécu les moments difficiles traversés par la Nouvelle-Calédonie durant la décennie Mais le choix des Calédoniens est d'aller aux urnes, et, encore une fois, nous avons grande confiance. L'essentiel, désormais, sera la nécessaire poursuite de la route commune, après le référendum. Les trente années qu'on a voulu être celles du rééquilibrage et de la construction d'un destin commun n'ont pas donné satisfaction à tous. Les jugements reflètent les clivages traditionnels : les uns en font trop, les autres, pas assez. années suffisent-elles pour atteindre de telles ambitions, de telles aspirations ? Ce sont des modes de vie, des cultures qui se sont engagés à dialoguer et à partager afin de se construire un destin commun. C'est un pari difficile, pour lequel il faut des acteurs humbles, respectueux de l'autre, honnêtes dans le constat et dans la poursuite des nouveaux objectifs à fixer. Je salue mes concitoyens originaires de Wallis-et-Futuna qui habitent en Nouvelle-Calédonie, où ils sont nombreux- près de 10 % de la population vivant sur ce territoire. Je les encourage à participer toujours avec ardeur, et dans le respect des autres, à la construction de leur terre d'accueil. terre d'accueil. À travers Pierre Frogier et Gérard Poadja, je souhaite à tous les responsables politiques, coutumiers, religieux, administratifs et associatifs de cette belle contrée du Pacifique, à laquelle je suis si attaché, courage et succès dans la préparation du référendum. À tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur origine, je veux redire

le climat doit être apaisé dès aujourd'hui. Les débats qui se déroulent sur le terrain, animés par le Haut-commissaire et à notre demande, ont pour objet de partager tout ce qui tout ce qui rassemble les Calédoniens, tout ce qui fait la force du dispositif qui se développe depuis trente ans. Ni plus, ni moins. Il en va de même pour la notion de peuple.

Michel Rocard. Mes chers collègues, il y avait tellement de violence, tellement d'incompréhensions, tellement de refus de se parler qu'il a fallu que quelqu'un adoptât dans la sphère politique une démarche inédite-

mais il a montré le chemin de la paix. Ce que Michel Rocard et de nombreux autres, des Calédoniens de part et d'autre, construisent depuis trente ans- on a, oui, donné du temps au temps, comme disait un Président de la République auquel Michel Rocard s'est parfois opposé

M. Stéphane Artano. Pour les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de Bélep, Lifou, Maré et Ouvéa, situées sur des îles environnantes, et de l'île des Pins, mais résidant en réalité à Nouméa, le projet de loi organique prévoit un droit d'option leur permettant d'exercer exceptionnellement leur droit de vote dans cette dernière Nous saluons ce dispositif, qui devrait permettre d'éviter des difficultés liées à l'exercice du droit de vote par procuration. Il devrait améliorer l'accès réel aux urnes des Néo-Calédoniens appelés à se prononcer sur un sujet aussi important. Toutefois, il importe de prendre en compte très en amont les complications qui pourraient surgir lors de l'application d'un dispositif à ce point dérogatoire, au risque d'altérer la légitimité de la consultation. Pour cela, les électeurs concernés doivent être très largement informés des modalités d'exercice de ce droit d'option et de son articulation avec la procuration, et cela le plus tôt possible, afin de dissiper toute ambiguïté. Compte Compte tenu des délais particulièrement resserrés que le Conseil d'État a relevés, nous avons jugé utile de prévoir un délai incompressible d'information des électeurs d'un mois avant la tenue de la consultation, afin que cette nécessité concrète soit bien prise en compte par le Gouvernement lorsqu'il prendra les mesures réglementaires nécessaires.

par avance toutes les dispositions d'information nécessaires, vous pourrez retirer vos amendements, parce que vous aurez toutes les garanties que vous en attendez. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Je veux parler des dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques, notamment la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, récemment enrichie par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, ou encore des dispositions pénales du code électoral qui prévoient des sanctions lourdes pour quiconque tenterait d'influencer le vote en s'appuyant sur ses moyens financiers.

d'avoir compris la responsabilité qui est la nôtre de contribuer à la création des conditions d'un scrutin incontestable en Nouvelle-Calédonie. Je crois que nous avons fait cette démonstration dans les meilleures conditions.

: Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 265, 2017-2018). Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (n° 105,